et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, inscrit à l'ordre du jour du mercredi 22 juillet 2020 après-midi, soit examiné selon la procédure normale et non selon la procédure simplifiée. Acte est donné de cette demande.

On parle fiscalité : notre fiscalité doit être remise en question. Les orientations européennes doivent être remises en question.

le défendre. Il vise à réduire de 20 % à 5,5 % le taux de TVA sur les prestations de réparation, afin d'enclencher une baisse de tarifs suffisamment incitative pour éviter le remplacement systématique des objets et prévenir le gaspillage.

qui limite l'application d'une TVA réduite à la réparation des vélos, chaussures, articles en cuir et linge de maison. Une extension à l'électroménager et aux équipements électriques et électroniques est à la fois logique et indispensable pour favoriser l'économie circulaire

bien mieux que moi. Nous proposons tout simplement d'appliquer un taux réduit de TVA à l'achat de bois labellisé ou certifié pour attester de son caractère local et durable.

Afin de garantir à nos concitoyens l'utilisation de bois en provenance de forêts exploitées durablement et de favoriser la relance économique de la foresterie locale et nationale, il convient d'appliquer le taux réduit de TVA à tout achat de bois labellisé ou certifié, ce qui atteste de son caractère local et durable. Soutenir l'achat d'un tel bois permet de favoriser une gestion forestière durable, c'est-à-dire écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable, selon la définition qui en qui en a été donnée au Sommet de la Terre, à Rio, en 1992. Une telle mesure permet également à l'État de soutenir la filière bois et forêts, qui fait actuellement face à une crise économique et sanitaire, liée non seulement à l'épidémie de covid-19, mais également aux scolytes, qui ont fortement impacté les finances communales dépendantes de ce secteur économique. Les auteurs de cet amendement souhaitent non seulement favoriser le bois durable, mais également le bois produit localement. Une telle démarche permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports des bois importés, d'introduire des circuits courts en limitant le nombre d'intermédiaires et de dynamiser le développement économique des filières de bois locales en provenance de forêts françaises. La parole

correspondant à la différence entre le prix de vente du bien et son prix d'acquisition initiale -, plutôt qu'à une TVA sur prix de vente, pour les ventes de terrains à bâtir intervenant dans le cadre d'opérations d'aménagement. Malheureusement, la doctrine fiscale a ajouté une condition, considérant que la TVA sur marge ne s'applique que lorsque la qualification juridique des biens n'est pas modifiée entre leur acquisition initiale et leur revente. Cette condition constitue un frein considérable pour tout projet d'aménagement, à l'encontre des politiques mises en place pour favoriser l'accès au logement. L'élargissement du périmètre de la TVA sur prix risque, dans les faits, de renchérir les prix du foncier et de rendre frileux les acteurs d'opérations d'aménagement. De plus, cette mesure constitue un facteur de baisse des droits de mutation perçus par les départements et les communes, dans la mesure où la TVA sur prix implique le paiement de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) à taux réduit, au lieu des DMTO dus à taux plein pour les opérations soumises à la TVA sur marge. Dans le secteur de l'aménagement, les collectivités locales ayant un rôle actif à jouer en faveur de la reprise économique, tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour conforter ce rôle. C'est dans cette perspective que le présent amendement tend à revenir à une application large de la TVA sur marge, conformément aux dispositions adoptées par le législateur en 2010, en prévoyant explicitement que le régime fiscal appliqué lors de l'acquisition initiale

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

Cette mesure simple, efficace, clairement identifiée par les ménages sera de nature à relancer l'activité des entreprises artisanales du bâtiment. Elle contribuera surtout à redonner du pouvoir d'achat aux particuliers qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation de leur logement. Le taux de TVA de 5,5 % a été appliqué dans le secteur du bâtiment de 1999 à 2011 et a permis de créer 53 000 emplois en soutenant l'activité de la filière. Comme pour le dispositif mis en oeuvre au travers de la dernière loi de finances rectificative pour 2020 pour l'application de la TVA à taux minoré aux masques

Le secteur du BTP a établi un guide de préconisations, validé par les ministères de la santé et du travail, en vue de permettre une reprise progressive des chantiers tout en assurant la sécurité des salariés. Cependant, ces mesures, qui sont laissées à l'appréciation de chaque entrepreneur, n'ont pu s'appliquer partout. Lorsqu'elles le sont, elles entraînent un surcoût important pour les TPE-PME. À la baisse de productivité résultant des surcoûts liés à la mise en place des protocoles sanitaires dans les entreprises est venue s'ajouter la majoration du coût de certains matériaux en raison des difficultés d'approvisionnement. Cette situation pose des difficultés pour les chantiers en cours ou les marchés signés. Une plus juste répartition des surcoûts entre les fournisseurs, les entreprises du BTP et les maîtres d'ouvrage

Les professionnels plaident pour qu'une ordonnance propre à la commande privée soit prise rapidement, en concertation avec l'ensemble des acteurs, afin que ce secteur économique essentiel soit préservé et en mesure de reprendre un rythme d'activité

l'avis du Gouvernement ? La majoration temporaire de la prise en compte des esters méthyliques d'acides gras, dits « d'hiver », avec une comptabilisation pour 1,2 fois leur valeur réelle, participe d'une démarche d'adaptation du secteur à la crise qu'il rencontre.

cet amendement vise à exonérer les collectivités territoriales de la TGAP pour les déchets qui ont été envoyés en installations de traitement thermique ou de stockage en raison de la crise sanitaire et qui ne l'auraient pas été en temps normal,

ne supporteraient pas le tarif majoré, c'est-à-dire que l'incinération de déchets autres que ceux pour lesquels l'installation a été autorisée ne donne pas lieu à l'application de tarifs majorés, de manière à répondre à des difficultés ponctuelles. Par ailleurs, nous travaillons avec les professionnels et les administrations concernés

sont susceptibles d'entraîner une forte majoration de la TGAP : 152 euros par tonne pour le stockage et 125 euros par tonne pour l'incinération. Les collectivités territoriales risquent donc d'être lourdement sanctionnées pour les conséquences des mesures qu'elles ont été contraintes de prendre en raison de la crise sanitaire. Le Gouvernement, par l'intermédiaire de la ministre de la transition écologique et solidaire, qui était alors Élisabeth Borne, et de sa secrétaire d'État Brune Poirson avait annoncé que la pénalité de TGAP ne serait pas appliquée aux collectivités

veillé, par l'entremise d'Élisabeth Borne, alors ministre de la transition écologique, à ne pas appliquer un certain nombre de majorations lorsque les installations n'étaient pas utilisées pour traiter les déchets habituellement reçus. Sur l'ensemble de ces amendements relatifs à la TGAP, le Gouvernement considère qu'il est plus sage, à ce stade, d'en rester aux équilibres existants. Par conséquent, l'avis est défavorable.

% permettant de bénéficier d'une réfaction de TGAP. Pour éviter que les collectivités territoriales et les opérateurs qui exploitent ces installations ne soient pénalisés fiscalement

Nous travaillons actuellement avec les professionnels et les administrations concernées à la recherche de solutions réglementaires, et nous considérons qu'il n'y a pas lieu d'inscrire de telles dispositions dans la loi.

Cet amendement vise à permettre l'instauration d'un dispositif de suramortissement des biens acquis par les agriculteurs afin de réduire leur exposition aux risques climatiques ou sanitaires,

au détriment de leur compétitivité, le plus souvent sans prendre en compte les réalités de nos territoires, au changement par l'innovation. Des équipements, dont la mise en vente a débuté, permettent de réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques

de pratiquer un suramortissement à hauteur de 40 % de la valeur d'origine des biens, hors frais financiers.

Cela signifie que nos services ont d'ores et déjà indiqué aux collectivités territoriales la possibilité de prendre de telles délibérations. Par conséquent, une modification importante du périmètre de cet article risquerait de rendre caduques des délibérations prises par anticipation par les collectivités

depuis des mois. En effet, ils ont dû mettre en oeuvre des dispositifs nouveaux, tel le fonds de solidarité, travailler à des remboursements anticipés des crédits d'impôt et des créances des entreprises sur l'État ou les collectivités,

Enfin, le travail sur la fiscalité est une chaîne continue, avec des étapes qui se succèdent : les retards que nos services prendraient contre leur gré engendreraient des risques sur les dates de production d'un certain nombre de documents ; je pense notamment à l'état 1259, qui conditionne les opérations budgétaires de l'année suivante.

Ces amendements partent du même constat : il semble peu raisonnable de fixer au 31 juillet 2020 la date limite pour décider de dégrèvements de CFE.

Est-ce cela, votre projet de décentralisation ?

l'ensemble des services de l'État et des collectivités territoriales font au mieux. Le système de la contribution

un creusement de l'écart entre la fiscalité perçue au titre des avances par douzièmes et la recette réelle de fiscalité une fois la décision prise et appliquée.

de la rédaction actuelle de l'article, le dispositif ne concerne qu'un nombre limité de secteurs affectés par la crise sanitaire. Pourtant, de nombreuses entreprises qui ne relèvent pas des secteurs des secteurs en question ont également été impactées, au plan économique, par les mesures sanitaires, en cela qu'elles fournissent des biens ou effectuent des prestations de services à des entreprises qui, elles, relèvent effectivement de ces secteurs.

L'article 3 permet aux communes et aux EPCI d'octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, aux entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l'événementiel. Cependant, le secteur de l'automobile a lui aussi été particulièrement affecté par le ralentissement de

L'amendement n° 681 est retiré. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demi, afin de poursuivre l'examen de ce texte. Il n'y a pas d'observation ? ... Il en est ainsi décidé.

en permettant aux travailleurs non salariés de débloquer de manière anticipée une partie de l'épargne retraite constituée les contrats de plan d'épargne retraite populaire (PERP). En effet, dans sa rédaction actuelle, le dispositif de l'article 4 ne porte que sur les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » et les plans d'épargne retraite individuels. Or, certains travailleurs non salariés ont souscrit non pas un de ces contrats, mais un PERP.

? Par ce dispositif, le Gouvernement souhaite apporter une aide ciblée, exceptionnelle et temporaire aux travailleurs non salariés, qui n'ont pas pu bénéficier des mesures de chômage partiel, et éviter de porter une atteinte disproportionnée à l'épargne retraite en étendant le déblocage à d'autres produits. Cette épargne permet de préparer un complément de revenu pour la retraite et elle soutient le financement à long terme des entreprises dans une période où celles-ci en ont besoin. Nous considérons que les PERP peuvent être débloqués de manière anticipée dans des cas limitativement énumérés par la loi, qui correspondent aux accidents de la vie et aux difficultés économiques, comme pour les autres produits d'épargne retraite. Ils bénéficient de possibilités de déblocage complémentaires sous certaines conditions, que nous souhaitons préserver,

Cet amendement vise à étendre le champ du dispositif prévu à l'article 4 en autorisant, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l'épidémie de covid-19, l'ensemble des travailleurs qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l'état d'urgence sanitaire à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.

ou de jours de repos, en l'absence de CET, vers un plan d'épargne entreprise, à condition que ces sommes servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou de parts ou actions de fonds d'actionnariat. Pour les entreprises, ces transferts seraient exonérés de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dans la limite de vingt jours par an et, pour les salariés, ils seraient exonérés d'impôt sur le revenu

les produits correspondants ouvrent droit à une exonération d'impôt sur le revenu, sans limite. Ce régime est donc déjà très favorable. Nous considérons que l'exonération de ces versements comporterait un risque élevé d'effet d'aubaine, étant donné que les plans d'épargne entreprise prévoient une durée de blocage de cinq années seulement et que les facultés de déblocage anticipé sont plus favorables que pour le plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco), ce qui limite l'investissement dans l'épargne longue et favorise les optimisations.

Il faudrait peut-être prendre conscience de la réalité que vivent des millions de gens qui n'arrivent même plus à payer leur loyer et à nourrir correctement leurs enfants. Voilà la situation des salariés, de ceux qui travaillent ! Je ne parle même pas de ceux qui ne trouvent pas de travail ...